La situation atteint un seuil critique. Les réseaux se dégradent, des missions sont annulées, les temps d'attente sont interminables, les rames sont bondées et les usagers souffrent. Île-de-France Mobilités annonce une augmentation importante du passe Navigo, qui serait porté à 84 euros. Les ménages ne peuvent pas supporter des coûts supplémentaires pour un service dégradé. Si l'enjeu des transports franciliens est avant tout de la responsabilité de la région Île-de-France et de sa présidente Valérie Pécresse, l'État ne peut pas s'y soustraire. La région capitale accueille de nombreux événements économiques et touristiques, dont les jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Surtout, ce réseau comptabilise 12 millions de voyages quotidiens, notamment de personnes qui travaillent. Alors que la pollution atmosphérique s'aggrave et provoque 6 000 décès prématurés par an, ce qui a conduit à la condamnation de notre pays pour une insuffisance coupable, le soutien aux transports collectifs doit être inscrit dans les priorités. L'arrivée prochaine du Grand Paris Express déséquilibrera encore plus les budgets d'Île-de-France Mobilités. quelles mesures le Gouvernement entend-il proposer lors de la conférence de financement ? Retiendra-t-il la TVA à 5,5 % pour affirmer une priorité aux transports collectifs ? Quelles marges de manoeuvre est-il prêt à donner sur le versement mobilité à la région Île-de-France et aux autres autorités organisatrices de la mobilité ?

pratiqués chez nos voisins européens. C'est notamment le résultat d'un choix de politique publique avec une prise en charge importante des coûts par la collectivité. La TVA sur les transports publics est d'ailleurs déjà au taux réduit de 10 %. Abaisser la TVA à 5,5 %,

à une hausse du versement mobilité. Ce serait non seulement pénaliser le coût du travail, à rebours de la politique du Gouvernement, mais également nuire à l'attractivité de la région. Le Sénat lui-même a rejeté une d'augmentation qui a été proposée dans le cadre du PLF pour 2023. Je rappelle également que les entreprises contribuent déjà pour moitié à la couverture des dépenses d'exploitation en Île-de-France, en prenant notamment à leur charge la moitié du coût des abonnements de leurs salariés. En outre, les recettes du versement mobilité ont augmenté de 5 % par an depuis dix ans. De son côté, l'État n'a jamais ménagé son soutien pour garantir la continuité d'un service public essentiel aux Français. Île-de-France Mobilités a ainsi bénéficié, dans le cadre de la crise sanitaire, d'une aide de plus

ministre déléguée. Cette mesure forte a pour but de venir en aide aux usagers et d'accompagner la mise en oeuvre des améliorations nécessaires et attendues de la qualité de l'offre de transports. Madame

que d'autres pays européens ont adoptée : ce serait une mesure utile pour les autorités organisatrices afin d'améliorer le service aux usagers. Les usagers n'ont pas à combler le trou de 950 millions d'euros d'Île-de-France Mobilités. Le Gouvernement, après avoir été silencieux durant tout le débat budgétaire au Sénat,

en lui demandant de faire annoncer le nom des stations par les conducteurs. Il y a quelques jours, un habitant d'Indre-et-Loire me sollicitait sur ce même sujet pour sa petite-fille, non-voyante, qui prend le métro parisien quotidiennement pour se rendre à son lieu de stage. Elle doit compter le nombre de stations afin de ne pas rater son arrêt. Imaginez la panique pour une jeune fille de 18 ans, venant de province de surcroît, dans ce grand labyrinthe qu'est le métro parisien Quelle ne fut donc pas ma surprise de retrouver cette question écrite, vieille de trente-trois ans, sur un sujet qui n'a toujours pas été réglé ... Le Gouvernement a récemment nommé Jean Castex à la présidence de la RATP

de 2005, laquelle prévoit une exception pour les réseaux souterrains de transports ferroviaires et guidés existants au 12 février 2005, dont le métro historique parisien. Pour ce qui concerne l'Île-de-France, les mesures relatives à l'accessibilité des lignes du métro parisien relèvent en premier lieu de la compétence de l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilités, en lien avec l'opérateur, la RATP. Île-de-France Mobilités a approuvé son agenda d'accessibilité programmée en 2015. Tous les quais et toutes les salles d'échanges des stations du métro parisien sont déjà équipés d'annonces visuelles et sonores. S'agissant de l'annonce sonore de la prochaine station à bord, les lignes en sont progressivement dotées au gré du renouvellement de leur matériel roulant, coorganisé par Île-de-France Mobilités et la RATP. ce jour, les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13 et 14 sont déjà équipées d'annonces sonores automatiques. La ligne 11 en sera équipée à la mise en service des nouvelles rames en 2023. Ce sera ensuite le cas de la ligne 6 à partir de fin 2023, puis des lignes restantes- 7, 8, 10, 12, 3 et 7 -avec la mise en service du nouveau matériel roulant MF 19 de façon progressive entre 2025 et 2035.

le 27 novembre dernier, le chef de l'État a annoncé son ambition de voir créer une dizaine de réseaux express régionaux (RER) dans les métropoles de France. Cette ambition, nous la partageons, car elle est bénéfique à l'environnement comme aux salariés

Avec 6,5 millions d'habitants, la région des Hauts-de-France est parmi les plus peuplées du pays, l'agglomération de Lille concentrant à elle seule 1,5 million d'habitants. Surtout, des dizaines de milliers de personnes s'y rendent chaque jour, en grande partie depuis le bassin minier. Le projet de Réseau express Grand Lille défendu par l'ancien conseil régional Nord-Pas-de-Calais devait permettre le désengorgement des accès à la métropole, mais il a été remisé à la faveur de la fusion des régions. Il prévoyait la création de six nouvelles gares, dont une gare souterraine

tous bords politiques confondus, à demander régulièrement la relance de ce projet. Aujourd'hui, à l'aune des annonces du Président de la République, il est temps de ressortir ce projet des cartons. Quels moyens seront alloués à la région Hauts-de-France pour ce projet, madame la ministre ? À quelle échéance les premiers voyageurs pourront-ils emprunter ces trajets ? La parole est à Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice

par l'amélioration des infrastructures des principales étoiles ferroviaires, de fournir une meilleure offre ferroviaire dans les grandes métropoles. En cohérence avec la priorité donnée aux mobilités du quotidien, au premier rang desquelles, vous l'avez dit, les relations domicile-travail, le Gouvernement soutient cette démarche aux côtés des collectivités concernées- régions et métropoles. À sa demande, SNCF Réseau a ainsi établi en 2020 un schéma directeur du développement des RER métropolitains. Par ailleurs, une enveloppe de 30 millions d'euros a été dédiée, dans le plan de relance, au lancement d'études de RER métropolitains dans les métropoles à fort potentiel, dont celle de Lille a été mise en place au cours des exercices 2021 et 2022. L'État finance ainsi, aux côtés de la région Hauts-de-France et de la métropole de Lille, les études de faisabilité lancées en 2021 visant à définir, puis à approfondir, un scénario de RER métropolitain pour l'étoile ferroviaire lilloise. Ce projet de grande ampleur, estimé à ce jour entre 4 milliards et 5 milliards d'euros, comprend- vous l'avez mentionné -un projet de barreau nouveau dénommé Réseau express Hauts-de-France entre Lille et le bassin minier. Comme le Président de la République l'a annoncé en février 2022, l'État sera présent aux côtés des acteurs locaux pour la mise en place de ce projet. La parole est à M. Patrice Joly,

des points de crispation demeurent tant sur la méthode employée que sur le fond du dispositif. Le Gouvernement a confié aux régions le soin de mettre en oeuvre cette nouvelle règle d'urbanisme ; son niveau de gestion réduit considérablement le rôle des élus locaux qui deviennent ainsi de simples exécutants devant se conformer à l'interprétation contraignante des règles. Je partage leurs inquiétudes de se voir déposséder d'une telle mission dans la gestion des espaces à aménager, alors même que ces élus de proximité, proches du terrain, disposent d'une connaissance fine des réalités locales et de leurs enjeux. Car le coeur du problème se trouve au niveau communal : comment justifier que des communes rurales soient évincées de la démarche, alors même qu'elles ont été, par le passé, peu consommatrices de foncier, qu'elles doivent faire face à l'accueil de nouvelles populations et travailler au développement de leur territoire ? Sur le déploiement et la temporalité du dispositif, il y a lieu de noter les délais fixés, relativement contraints, qui ne laissent pas suffisamment de place au dialogue, à l'interaction et à la coconstruction. En effet, le conseil régional assure le pilotage du ZAN avec comme principal interlocuteur la conférence des

ruraux, pouvez-vous m'indiquer les garanties que vous comptez apporter à des territoires peu consommateurs de foncier par le passé afin qu'ils puissent bénéficier du foncier nécessaire à leur développement et à l'accueil de populations ? Quels aménagements entendez-vous mettre en oeuvre pour que la réalisation de cet objectif puisse se concrétiser sans pénaliser les territoires ruraux ? Enfin, avec mes collègues du groupe socialiste, nous nous sommes positionnés en faveur du report de la première étape de réalisation de l'objectif fixé à 2030. Quelle est votre position quant à cette demande ? La parole

il m'a chargée de vous répondre. Chaque année, ce sont en moyenne 20 000 hectares d'espaces agricoles, naturels et forestiers qui sont consommés en France. La lutte contre l'artificialisation est un enjeu majeur pour préserver les sols, la biodiversité et l'activité agricole. La France s'est donc fixé l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050 avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années, donc à l'horizon 2030, comme vous l'avez indiqué. Tous les territoires sont concernés, y compris les territoires ruraux. Sur la dernière décennie, la consommation d'espaces est d'ailleurs majoritairement, à hauteur de 61 %, localisée sur les territoires détendus, plus particulièrement en périurbain peu dense à très peu dense. Tous les territoires doivent donc contribuer à l'atteinte de cet objectif, même si la loi prévoit que leur effort sera modulé en fonction de leurs besoins spécifiques. Cette trajectoire progressive est à décliner dans les documents de planification et d'urbanisme

à l'ordre du jour. La territorialisation de la trajectoire ZAN devra moduler le rythme d'artificialisation des sols en tenant compte des besoins et des enjeux locaux : dynamiques démographiques et économiques, équilibre du territoire. Cette dernière dimension comprend la question du désenclavement rural, et il est clair que nous pourrons donc continuer à construire dans ces territoires. Néanmoins, et pour rassurer les élus quant à la bonne prise en compte de cet enjeu, la Première ministre, en clôture du Congrès des maires, a formulé plusieurs annonces dans le prolongement de discussions que nous avons eues avec les associations d'élus et les parlementaires. Elle s'est notamment engagée à étudier des pistes en vue de garantir que toutes les communes rurales puissent bénéficier de possibilités de construction, en particulier lorsqu'elles ont peu construit par le passé. Elle s'est aussi engagée à permettre la contractualisation entre l'État et le bloc communal en cas de blocage au niveau des territoires pour trouver des solutions et parvenir à un équilibre entre développement de projets d'intérêt majeur et sobriété foncière.

Avec l'augmentation des grands projets urbains, les espaces naturels et les terres agricoles sont devenus autant de décharges potentielles pour certaines grandes entreprises du bâtiment, lesquelles n'hésitent pas à contourner les règles pour y déverser leurs tonnes tonnes de gravats, dont certains peuvent s'avérer dangereux. Ayant été interpellée à plusieurs reprises par les élus locaux et les acteurs associatifs, je partage pleinement leurs préoccupations relatives aux questions environnementales et à la dégradation du cadre de vie des habitants des villes moyennes, des petites villes et des villages situés à la périphérie des grandes métropoles. Je comprends parfaitement leur profond sentiment d'injustice face à l'absence de réaction étatique. Il est primordial de conserver la biodiversité de l'environnement des communes de la grande couronne parisienne dans un esprit d'égalité des territoires. Aussi, il est urgent d'apporter des solutions immédiates, particulièrement pour les communes de Fleury-Mérogis, Cheptainville-Lardy et Saint-Hilaire, qui sont démunies face à ce phénomène et qui ont besoin d'aide pour réhabiliter leurs terrains et espaces naturels pollués par ces exhaussements, dits aussi remodelages. Nos villes et villages n'ont pas vocation à devenir les victimes collatérales du développement urbain des métropoles et grandes agglomérations. Il s'agit d'une inégalité environnementale manifeste, qui s'ajoute, dans un silence inadmissible, aux inégalités sociales et territoriales déjà bien ancrées dans ce département. Je souhaiterais connaître, madame la ministre, les mesures que vous envisagez de prendre pour protéger les territoires essonniens contre ces atteintes graves à l'environnement qui ont un impact sur la vie quotidienne des habitants. Il est temps de se saisir de cette question sensible et importante un terme à ces pratiques scandaleuses, totalement en contradiction avec les engagements issus de la Convention citoyenne pour le climat. La parole

en Essonne et leur impact environnemental et agricole. Tout d'abord, je rappelle que les installations de stockage de déchets inertes sont des équipements importants pour la protection de l'environnement. Elles permettent d'éviter que des terres excavées ou certains déchets de chantiers ne soient dispersés dans l'environnement, sous forme de dépôts sauvages, et garantissent que le stockage est réalisé dans des conditions respectueuses de l'environnement. Les conseils régionaux sont responsables la planification de ces installations de stockage. Les services de l'État chargés de l'environnement s'assurent que ces installations soient implantées et exploitées dans de bonnes conditions de sécurité et de respect de l'environnement, notamment au titre de leurs missions d'instruction et d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. En ce qui concerne les trois projets que vous évoquez, les situations sont différentes. Dans le cas de Saint-Hilaire, un projet d'installation de stockage était effectivement prévu. Néanmoins, une instance de classement au titre des paysages ayant été signée par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la procédure d'autorisation environnementale est suspendue, rendant l'avenir du projet incertain. Dans le cas de Fleury-Mérogis, il s'agit non pas d'un projet d'installation de stockage, mais d'un programme d'aménagement agricole et de mise en culture réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la commune et sur des terrains lui appartenant. Enfin, dans le cas de Cheptainville-Lardy, si la commune a été approchée sur le sujet, il n'y a, à ce jour, aucun projet d'installation de stockage déposé auprès des services de l'État. En tout état de cause, la création d'installations de stockage en Île-de-France répond à un réel besoin, identifié dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets d'Île-de-France. Celui-ci fait en effet état de la nécessité de créer de nouvelles capacités de stockage de terres, à hauteur de 2 millions de tonnes par an jusqu'en 2025. Par ailleurs, ce plan encourage le rééquilibrage territorial des capacités de stockage de déchets inertes vers l'ouest et le sud de la région Île-de-France, la Seine-et-Marne accueillant actuellement environ 70 % du tonnage régional de déchets inertes. La parole

de pertes ovines possiblement imputables au loup le plus élevé, mais c'est aussi le pays dont les aides publiques à la protection et à l'indemnisation des troupeaux sont les plus élevées eu égard au nombre de loups. Deux hypothèses : soit Deux hypothèses : soit le nombre de pertes ovines possiblement dues aux loups est surestimé, soit la protection des troupeaux est inefficace, voire non effective. Ainsi, M. Bazin souhaiterait connaître : les critères permettant d'attribuer les pertes au loup loup ; le pourcentage de relevés techniques réalisés sur le lieu de l'attaque rapporté au nombre de constats déclaratifs ; et, enfin, le nombre de comptes rendus de visites et contrôles sur place, de contrôles de schéma de protection et du cahier de pâturage, effectués et analysés par les services instructeurs. La Commission européenne, dans la communication précitée, estime que le système français est un bon exemple de système de surveillance précis permettant d'obtenir des données solides et appropriées à la conservation et la gestion des loups.

Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur les raisons du niveau élevé de prédation par le loup en France, malgré le financement public considérable des moyens de protection des troupeaux. Cela s'explique à la fois par la présence d'un élevage pastoral avec des troupeaux parfois importants dans les zones de présence du loup, et par l'existence de nouvelles zones de prédation n'ayant pas fait encore l'objet de mesures de protection. Il est important de rappeler que la France est le seul pays où le coût du gardiennage est pris en charge par la collectivité. En ce qui concerne l'éventuelle surestimation du phénomène, il apparaît normal qu'en cas de doute sur l'attribution de la responsabilité d'un dommage à un prédateur, ce doute profite à l'éleveur. ailleurs, les constats déclaratifs restent aujourd'hui très minoritaires par rapport à ceux réalisés par des agents publics. Ils sont réservés aux troupeaux situés dans des départements de présence ancienne du loup, et aux cas d'attaques faisant moins de cinq victimes. En dehors des zones nouvelles de prédation, les indemnisations de dommages sont subordonnées à la mise en place de mesures de protection. Des efforts sont faits à cette fin, avec notamment une démarche engagée auprès des élevages subissant les plus fortes prédations. Inauguré en 2020, cet accompagnement concerne aujourd'hui les 200 élevages concentrant 50 % de la prédation. Cela alimente également l'observatoire des mesures de protection, qui est en cours de développement. La mise en oeuvre effective des mesures de protection est d'abord contrôlée dans le cadre de leur financement par l'État au titre de la bonne utilisation des fonds publics. Elle l'est également dans le cadre de l'instruction des demandes de tirs de défense, et, systématiquement, avant chaque tir effectué par les louvetiers ou la brigade d'intervention de l'OFB. d'intervention de l'OFB. La méthode française de suivi de la population de loups est reconnue comme l'une des plus complètes et efficaces en Europe. Il est en revanche essentiel que la confiance demeure entre tous les acteurs concernés, éleveurs comme comme chasseurs. Des efforts ont été entrepris en ce sens depuis la fin de l'année 2021. Ils ont porté leurs fruits, puisque davantage d'indices de présence ont été collectés au cours de l'hiver 2021-2022. Le fait que les tirs augmenteraient la prédation reste une hypothèse, ni confirmée ni infirmée. Des recherches sont encore en cours à ce sujet. En tout état de cause, depuis quelques années, priorité est donnée aux tirs de défense effectués sur des loups en situation d'attaque.

Entre les rattrapages de charges de l'année 2021-2022 et les appels de charges pour 2023, bon nombre de copropriétaires sont aujourd'hui pris en étau, avec le risque d'une multiplication des défauts de paiement, voire d'abandon de projets de travaux de rénovation énergétique, ce qui est pour le moins paradoxal. Le bouclier tarifaire présente aujourd'hui deux problèmes majeurs. Tout d'abord, il n'est compensé qu'après les avances de charges, courir un reste à charge exorbitant le temps de sa mise en oeuvre. Ensuite, il est très nettement sous-dimensionné au vu de l'explosion du prix du gaz et de la hausse des factures. Par exemple, dans une copropriété comme celle du Parc Lubonis à Nice, le devis pour les charges de chauffage s'élève à plus de 600 000 euros, le bouclier tarifaire s'appliquant à hauteur de seulement 91 076 euros. 91 076 euros. Le reste à charge serait donc de 593 703 euros, soit une augmentation des frais pour les copropriétaires de 593 % ! Résultat : le conseil syndical a décidé de ne pas mettre en route le chauffage collectif. Combien de temps cela pourra-t-il durer avec l'arrivée du grand froid ? Madame la ministre,

des TRV hors gel. Le ministre de la ville et du logement et la ministre de la transition énergétique sont pleinement mobilisés pour assurer une égalité de traitement entre tous. Parce que nous devons aller vite, le texte couvrant le deuxième semestre 2023 est sorti le 15 novembre dernier, pour apporter une réponse dès que possible. Le Gouvernement est également engagé dans la mise en place d'une aide pour les contrats signés dans des conditions très très défavorables, et qui ne sont pas bien couverts par le bouclier. S'agissant du décalage entre les versements et les besoins en trésorerie, la loi de finances pour 2023 va permettre aux copropriétés disposant d'un contrat de fourniture de gaz de bénéficier du versement de l'aide équivalente aux boucliers directement sur leur facture. Si cela ne répond pas à toutes les situations, nous envisagerons alors une aide spécifique pour répondre aux besoins de trésorerie, et éviter ainsi de laisser des copropriétés en difficulté dans l'attente du versement de l'aide bouclier. Vous pouvez être assurée, madame la sénatrice, de l'entière

Présenté dans le cadre des Assises nationales du transport aérien en 2021, ce concept vise à réduire les nuisances sonores des aéronefs commerciaux amorçant leur descente lorsqu'ils sont à proximité des habitations et lorsque leur plan de vol ne permet pas d'autre itinéraire. Depuis 2016, cette procédure est parfois utilisée pour les vols de nuit ou pendant les périodes de moindre trafic. Sa généralisation ne serait certes pas sans conséquence sur l'organisation des flux aériens dans le ciel francilien, mais la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) prévoit bien un déploiement opérationnel du concept à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle à l'horizon 2023. Pour de nombreux vols, et particulièrement les vols transatlantiques, la descente vers l'aéroport de Roissy commence dans le ciel yvelinois, ou du moins dans les départements de l'ouest francilien. Beaucoup de communes des Yvelines subissent donc d'insupportables nuisances sonores, nocturnes et diurnes, dues au trafic aérien. L'hypothèse d'une réduction du bruit est scrutée avec attention et impatience par nos concitoyens et par les élus locaux de ces territoires. La DSNA l'a confirmé, après son annonce par la précédente ministre des transports, Mme Borne, la généralisation des descentes douces serait pour 2023. Madame la ministre, alors que nous approchons à grands pas de la date butoir sans pour autant être informés d'évolutions imminentes,

nuisances sonores des aéronefs commerciaux à destination de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. La descente douce ou descente continue est une technique de pilotage qui permet l'optimisation des profils verticaux de descente par les pilotes, et ce grâce à des procédures de circulation aérienne adaptées et basées sur des données de positionnement par satellite. Dans la continuité des annonces faites à l'occasion des Assises nationales du transport aérien, des études techniques et opérationnelles de conception de telles procédures ont été lancées par la Elles ont conduit à la réalisation de tests grandeur nature sur une des pistes d'atterrissage de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Ces expérimentations ont été mises à profit pour analyser les impacts opérationnels, environnementaux réglementaires de telles procédures, dans le contexte très spécifique de cet aéroport doté de quatre pistes exploitées simultanément. Les travaux techniques sont toujours en cours. Ils concernent notamment la définition des procédures d'approche, leur exploitation par les pilotes, l'analyse des éventuels impacts sur la sécurité des vols et, enfin, les les conséquences sur les conditions de survol des territoires potentiellement concernés par ces changements. Un calendrier précis pourra être élaboré et proposé aux parties prenantes lorsque ces études parviendront à leur terme. Le projet de mise en service de descentes douces à Paris-Charles-de-Gaulle sera bien entendu présenté aux instances de concertation. Il fera, selon toute vraisemblance, l'objet de l'organisation d'un débat public par la Commission nationale du débat public (CNDP),

Cette situation devrait aller en s'aggravant en 2023 en raison de la hausse du prix de l'électricité pour les parties communes et de celle du gaz pour les chaufferies collectives, prévues dès le mois de janvier 2023. Dans mon département d'Indre-et-Loire, cette situation a conduit de nombreux locataires à manifester contre l'augmentation des charges communes, ce qui a contraint certains offices publics de l'habitat à procéder à un lissage des charges locatives. Le delta facturé aux locataires des parcs sociaux restant élevé en dépit des mesures prises par le Gouvernement, le nombre des impayés devrait considérablement augmenter dans les mois qui viennent. Aussi, je souhaiterais savoir si, et dans quelle mesure, le bouclier énergétique pourrait être plus favorable aux locataires du parc social, et si les bailleurs sociaux pourraient bénéficier du bouclier tarifaire pour leur consommation d'électricité dans les parties communes.

Les bailleurs sociaux du département sont extrêmement inquiets. Madame la ministre, avez-vous connaissance de ces difficultés ? Quelles sont les solutions envisagées ? La parole

aux ménages chauffés collectivement au gaz naturel ou par un réseau de chaleur utilisant le gaz naturel. Comme pour les tarifs réglementés, ce bouclier a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Un décret, publié le 15 novembre dernier, précise ainsi les modalités pratiques de cette prolongation. Un autre décret, en cours de concertation, étendra prochainement le bouclier tarifaire aux ménages bénéficiant d'un chauffage collectif électrique. Ce bouclier sera rétroactif à partir du mois de juillet, et étendu sur toute l'année 2023. Le périmètre permettra une couverture de tous les logements, y compris les logements du parc social, ainsi que des parties communes. L'objectif du Gouvernement est évidemment de protéger tous les Français de la même manière. Nous travaillons d'ailleurs très étroitement avec l'ensemble des acteurs pour veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. Par ailleurs, s'agissant du chèque énergie, nous mènerons des travaux complémentaires pour déterminer comment les locataires de logements dotés d'un chauffage collectif pourraient utiliser ce chèque pour régler directement leurs charges, ce qui pose aujourd'hui des difficultés juridiques et opérationnelles. Dans l'attente de ces travaux, je souhaite insister sur le fait que ces locataires peuvent d'ores et déjà utiliser le chèque énergie dont ils sont bénéficiaires pour le paiement de leur facture d'électricité individuelle, liée à leur propre contrat. La parole

? En cas de débordement des eaux usées ou d'arrêt du fonctionnement des stations de pompage ou d'épuration, qui ne peuvent pas toutes disposer de groupes électrogènes, on encourt en effet des risques importants en matière d'alimentation

d'assainissement collectif. Il est tout à fait incompréhensible que les services publics de l'eau et de l'assainissement ne constituent pas, de façon systématique, des activités relevant des services prioritaires, au vu des incidences en termes de salubrité publique et de pollution. alors que des aides de compensation sont prévues pour les entreprises du secteur de l'eau et de l'assainissement de droit privé, les régies publiques du même secteur n'y seraient pas éligibles. En Charente-Maritime, la régie d'exploitation des services d'eau est le premier opérateur de production et de distribution d'eau potable sous statut d'établissement public à caractère industriel et commercial ; ses dépenses d'électricité devraient passer de

sa plus grave crise énergétique depuis les chocs pétroliers des années 1970. La crise ukrainienne et la volonté de la Russie d'utiliser l'approvisionnement énergétique comme moyen de pression entraînent des tensions sans précédent sur les marchés du gaz et, par voie de conséquence, sur les marchés électriques. La communication réalisée par le Gouvernement depuis la fin du mois de novembre a permis de rappeler que toutes les dispositions nécessaires pour aborder l'hiver dans les meilleures conditions possible ont été prises ou sont en cours d'instruction. Le premier levier activé est celui de la réduction de notre consommation d'électricité, qui s'intègre dans la démarche plus globale du plan de sobriété énergétique. Le second levier est celui de la maximisation des moyens de production. Cela passe d'abord par le suivi rapproché de la disponibilité de la disponibilité nucléaire et par la sécurisation de nos approvisionnements en gaz. Cela passe aussi par l'accélération des projets d'énergies renouvelables en cours ou par l'autorisation d'usages à des seuils supérieurs au cadre usuel. que, si le système électrique venait à être confronté à une situation de tension inédite et si tous les autres leviers activés se révélaient insuffisants, des coupures des coupures locales, ciblées et temporaires pourraient théoriquement intervenir en dernier recours pour certains usagers raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité. Les installations d'eau potable et d'assainissement ne figurent pas explicitement dans l'arrêté du 5 juillet 1990 fixant les catégories d'usagers dits « prioritaires ».

prioritaires, le Gouvernement a conscience du besoin de réinterroger les critères de priorité inscrits dans l'arrêté du 5 juillet 1990. Dans le cas où des évolutions seraient nécessaires, celles-ci ne devraient toutefois pas conduire à élargir trop sensiblement le champ des usagers pouvant être priorisés, car les consommations électriques préservées ne doivent pas dépasser 38 % de la consommation du département. Ce travail pourra être mené en 2023, à l'aune du retour d'expérience de l'hiver 2022-2023. La parole

de la région ont relevé un nombre important d'éoliennes défectueuses, notamment sur le site de Widehem. Je me suis rendue sur place pour constater qu'effectivement de nombreux moulins ne tournaient pas, ou ne tournaient Les pales étaient, pour la plupart, manquantes ou cassées. Ces éoliennes avaient été mises en service en 2000 et 2001. Or la tempête du 6 janvier 2012 a déchiqueté les pales de nombreuses installations. aucune réparation n'a été constatée jusqu'à présent. Chaque élu cherche à lutter contre la pénurie d'énergie qui frappe notre pays. Il nous faut cependant préserver nos sites naturels d'une pollution visuelle et terrestre, en obligeant les

La crise actuelle nous rappelle l'importance de la maîtrise de notre production d'énergie. Nous devons mettre fin à notre dépendance énergétique vis-à-vis d'autres pays. C'est pourquoi le Gouvernement agit pour accélérer le développement des énergies non carbonées, à savoir les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire.

de l'État pour accélérer le traitement des projets. Le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables constitue le volet législatif de ce grand plan.

au projet initial ». Il est donc légitime de s'interroger sur l'utilisation la plus efficiente possible des éoliennes et sur la manière dont elles peuvent être réparées ou démantelées. Le cadre réglementaire actuellement en vigueur se fonde sur l'arrêté ministériel du 26 août 2011, qui a été modifié le 10 décembre 2021

Cet accord devrait donner lieu à un règlement européen dans les toutes prochaines semaines. La parole

Dans le cas des élections sénatoriales des Français établis hors de France, l'atteinte que porte le vote par procuration au principe de secret du suffrage est plus que légitime et légitime et proportionnée. L'article 53 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France permet le vote par procuration. Son article 51 exige que la liste d'émargement reste déposée sur la table du bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote, mais ne prévoit nullement que ce registre doive être communiqué avant le vote. Pourtant, le secrétariat de l'Assemblée des communique aux membres du collège électoral qui en font la demande le registre des procurations, avant le vote. Ce registre dématérialisé, facilement communicable à des tiers, contient les noms des mandants et de leurs mandataires.

À ce titre, il fait l'objet d'une procédure encadrée et contrôlée, en particulier pour éviter toute fraude électorale. Dans ce cadre, seul le registre des procurations permet à un électeur doutant de la régularité de l'établissement d'une procuration de soulever ce grief à l'appui d'une saisine du juge électoral. Afin de garantir l'effectivité du contrôle des procurations par les électeurs, ce registre, désormais extrait du répertoire électoral unique (REU), comprend toujours les noms et prénoms du mandant et du mandataire, ainsi que l'identité et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration, la date et le lieu de son établissement, et la durée de validité de la procuration. Ces éléments sont des garanties tant pour les électeurs qui souhaiteraient introduire un recours que pour les membres du bureau de vote, car ils leur permettent de contrôler la véracité des procurations et ainsi la transparence et la sincérité du scrutin. Le registre est un instrument indispensable pour examiner à la fois les identités des mandants et des mandataires et le respect du plafond des procurations. Dès lors, la mise à disposition du registre des procurations, même dans le cas que vous évoquez d'un collège électoral peu nombreux, est indispensable. Néanmoins, pour répondre précisément à votre interrogation, le seul fait de pouvoir identifier le mandant et le mandataire d'une procuration sur le registre des procurations ne saurait constituer une atteinte au secret du vote, dans la mesure où cette identification ne conduit pas à une divulgation réelle du choix de l'électeur. Si un électeur se trouvait être soumis à des pressions, il devrait saisir sans attendre le juge électoral, qui est compétent pour rechercher si d'éventuelles manoeuvres ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. C'est pour ces raisons, madame la sénatrice, que le Gouvernement n'envisage pas de supprimer les mentions relatives aux noms et prénoms des mandataires sur le registre des procurations. La parole

Il se révèle vital pour ceux qui résident dans des zones rurales ou périurbaines, là où les Français ne peuvent compter que sur des solutions de transport personnelles pour leur vie sociale, scolaire et professionnelle. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une double réalité : d'un côté, les mesures mises en place pour faire baisser le prix du permis de conduire ne sont pas suffisamment opérantes ; de l'autre, les écoles de conduite voient leurs frais augmenter drastiquement du fait de l'inflation. Seule une action concrète sur les financements permettrait d'aider les jeunes à accéder à la mobilité et à l'emploi. Les professionnels proposent de mettre en oeuvre une mesure utile, qui profiterait à la grande majorité des jeunes et aurait un impact financier limité pour l'État l'État : la portabilité du compte personnel de formation (CPF) au sein de la cellule familiale. Ainsi, les parents pourraient utiliser tout ou partie des sommes créditées sur leur compte personnel de formation pour financer la formation de leurs enfants au permis de conduire.

En effet, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a instauré un droit individuel utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, y compris en période de recherche d'emploi, pour suivre une formation certifiante.

L'initiative que vous proposez pourrait être intéressante, mais les droits au CPF reposent sur cette contribution qui vise à couvrir les demandes des bénéficiaires s'inscrivant dans une démarche individuelle de formation ; à ce titre, ils ne peuvent devenir cessibles. au permis de conduire est aujourd'hui une action éligible au CPF, dans la mesure où elle contribue à la réalisation ou à la sécurisation du projet professionnel du titulaire du compte. En outre, le Gouvernement a développé plusieurs aides afin d'accompagner les jeunes de 15 à 25 ans, les apprentis d'au moins 18 ans, les demandeurs d'emploi et les personnes en situation de handicap dans le financement de leur permis de conduire.

sa dernière demeure. Une forêt cinéraire est définie comme un site d'inhumation d'urnes funéraires biodégradables. Elle permet de vivre le deuil différemment, en offrant des lieux de mémoire et de recueillement en pleine nature,

Malheureusement, dans notre pays, la réglementation peut être bloquante, comme a pu nous le montrer l'exemple de la commune d'Arbas, en Haute-Garonne, dont le projet a été arrêté en raison de blocages administratifs dus à des contradictions au sein des services de l'État. Ces contradictions résultent d'incompatibilités avec le droit funéraire en vigueur : en France, disperser les cendres d'un défunt en pleine nature

En Alsace, les communes sont de plus en plus nombreuses à vouloir disposer d'une forêt cinéraire et trouvent, à cette fin, d'autres solutions. C'est le cas de la commune de Muttersholtz,

La création et la gestion de ces sites reviennent exclusivement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les projets que vous évoquez ne peuvent être mis en oeuvre car ils sont incompatibles avec le droit funéraire en vigueur. En effet, l'inhumation d'une urne biodégradable dans ce type de site, après réservation d'un emplacement, revient à faire payer aux familles des prestations qui doivent être gratuites. En l'état actuel du droit, la dispersion des cendres à l'issue de la crémation est notamment autorisée « en pleine nature ». Cette opération, qui peut par exemple s'effectuer au sein d'un espace naturel forestier, est gratuite, mais ne peut donner lieu à la matérialisation d'une sépulture. Le Gouvernement reste toutefois attentif à cette situation et aux attentes des élus locaux souhaitant s'engager dans ces projets. Afin de les accompagner, les services de l'État demeurent à la disposition des collectivités qui souhaitent, dans le respect du droit en vigueur et en veillant à la protection des intérêts des familles et de la dignité des défunts, créer un site cinéraire isolé, à l'esthétique et au fonctionnement plus écologiques que les cimetières et les sites cinéraires traditionnels. La parole

L'acquisition de nouveaux appareils- deux en 2021 et deux en 2022 -a ainsi permis, dans un temps court, de résoudre en partie les difficultés liées aux défaillances du prestataire logistique et au vieillissement du parc

d'ouverture des bases et détachements existants en lien avec les ressources humaines disponibles. Une étude sur l'implantation et la répartition actuelle des bases pourra alors être conduite, en lien avec les implantations des hélicoptères de la gendarmerie nationale et de celles des HéliSmur du service mobile d'urgence et de réanimation (Smur). Elle concernera bien entendu la faisabilité de l'ouverture d'une base dans la zone de défense nord.

Ces implantations permettent donc de couvrir actuellement les besoins en l'absence d'hélicoptère de la sécurité civile. La parole

pour sanctionner le non-paiement du stationnement. Elle a conclu une convention avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai), qui est chargée de l'envoi du forfait de post-stationnement à l'adresse de la carte grise des propriétaires de véhicules en défaut de paiement. Si ce forfait de post-stationnement n'est pas acquitté dans les délais, la direction générale des finances publiques (DGFiP) adresse un avertissement avec une majoration

sur la preuve de l'envoi de ce forfait à l'adresse référencée sur la carte grise du requérant. L'Agence n'apportant jamais la preuve demandée, la CCSP annule systématiquement la majoration et demande à la collectivité d'adresser à l'Antai cette décision d'annulation.

Toutefois, la collectivité a constaté que la décision d'annulation n'est pas systématiquement transmise à la DGFiP, car les requérants qui n'ont pas obtenu remboursement sollicitent la CCSP pour faire exécuter les décisions. La collectivité regrette l'illisibilité du processus et craint donc que cela n'aboutisse à des condamnations pécuniaires à son encontre. Madame la secrétaire

L'Agence joue ainsi un rôle double : d'une part, elle assure, pour les collectivités qui en font le choix, l'édition et l'envoi des avis de paiement des forfaits de post-stationnement (FPS) ; d'autre part, elle émet le titre permettant la majoration de 50 euros pour le compte de l'État, si l'avis de paiement de FPS n'a pas été réglé dans un délai de trois mois. En 2021, l'Agence a ainsi adressé plus de 11 millions d'avis de paiement de FPS pour le compte de différentes collectivités locales, dont environ 132 000 pour la ville de Rouen-

Toutefois, la jurisprudence de cette juridiction administrative tend à ne pas reconnaître à ces informations la valeur de preuve de la notification. Afin de trouver une solution à ce problème, l'Agence développe, depuis 2021, une interconnexion informatique avec la CCSP qui devrait permettre, à terme, la transmission des éléments de preuve quant à la notification des avis de paiement de FPS. concerne les décisions rendues par la CCSP, et contrairement à ce qui a pu être indiqué, l'Antai transmet systématiquement à la DGFiP les messages d'annulation de FPS envoyés par les collectivités. Néanmoins, l'augmentation du nombre de requêtes déposées devant la CCSP au fil des ans-

et automatisé du remboursement à un traitement manuel qui allonge, par définition, les délais de remboursement. La parole

secrétaire d'État. Madame la sénatrice Vogel, le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) pour nos concitoyennes est l'un de nos droits fondamentaux les plus absolus. Nul- je dis bien nul -ne doit pouvoir retirer aux femmes le droit de disposer de leur corps. C'est pourquoi le Président de la République a annoncé, dès janvier dernier, vouloir l'inscrire dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision choquante et incompréhensible de la Cour suprême outre-Atlantique n'a fait que renforcer notre volonté Certains diront que l'exemple américain n'a pas sa place en France. Certes, nos institutions fonctionnent différemment ; le droit à l'IVG est ici mieux protégé. Mais, de grâce, ne prenons pas de risque, car il suffira d'une crise pour que le droit des femmes soit remis en cause ! C'est pourquoi, comme l'ont annoncé la Première ministre et le garde des sceaux, le Gouvernement appuiera toutes les initiatives parlementaires engagées sur cette question. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait le 19 octobre dernier en soutenant avec force votre proposition de loi, madame la sénatrice. Malheureusement, ce texte, qui évoquait également la contraception, a été rejeté de seulement 17 voix- nous le regrettons. Vous le savez, le 24 novembre dernier, le garde des sceaux a de nouveau répondu présent en soutenant la proposition de loi de la présidente Panot qui a, elle, été largement adoptée à l'Assemblée nationale, ce dont le Gouvernement se félicite. Je note d'ailleurs que, pour concentrer nos efforts, la majorité et la présidente Aurore Bergé ont retiré leur Il revient désormais au Sénat de se prononcer sur la nouvelle version adoptée, qui est selon nous plus à même de faire consensus en ce qu'elle ne mentionne pas la contraception et renvoie à la loi. En effet, je rappelle que, en matière de révision constitutionnelle,

la filière gras nage en plein cauchemar. Le 6 décembre, trois nouveaux foyers d'influenza aviaire ont été détectés en Dordogne. Quelque 600 éleveurs du Périgord sont menacés, et avec eux toute une économie basée sur la vente directe ou l'agrotourisme. L'activité des acteurs de la filière périgourdine a été réduite de 60 % du fait de la grippe aviaire, alors que la crise sanitaire avait déjà entraîné une mise à l'arrêt de la production. Plans de mise à l'abri, de claustration et d'abattage des bêtes ... Ces moyens de lutte contre la propagation de l'épidémie sont efficaces, mais ne doivent pas constituer la panacée. Il nous faut un vaccin, et vite ! Face aux pertes colossales engendrées par cette épidémie, nous devons impérativement soutenir la filière. Les éleveurs sont pris à la gorge. Certains n'ont pas encore reçu le solde des abattages d'avril et sont de nouveau contraints de réduire leur nombre d'animaux ... Il y a véritablement urgence. Pourtant, les aides et subventions de l'État ne sont pas à la hauteur. Dépenses de mise aux normes, achat de nouveaux animaux, frais énergétiques en hausse : la filière est plus que jamais fragilisée. Nous devons aller plus loin dans l'accompagnement des acteurs et dans la prise en charge totale des pertes, et ce dans des délais raisonnables. Monsieur le ministre, le 7 décembre, vous disiez ici même qu'une partie de la filière aurait disparu sans les aides accordées l'année dernière. Personne ne le conteste. Toutefois, la situation a encore empiré et rien ne présage une embellie. Envisagez-vous de renforcer les aides accordées à la filière ? Avez-vous des précisions à apporter aux éleveurs concernant le vaccin ?

de la souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre, j'ai été interpellée par les agriculteurs de la commune de Wambaix, dans le département du Nord, qui m'ont exposé la situation alarmante qu'ils connaissent en raison de la hausse des coûts de l'énergie. En effet, les plants de pommes de terre doivent être conservés dans des bâtiments frigorifiques à une température de 2 degrés, pendant plus de sept mois, avant d'être expédiés aux agriculteurs chargés de les planter. L'électricité est donc un facteur de production crucial pour la filière.

Malgré des travaux d'isolation, les factures pourraient atteindre jusqu'à 500 % d'augmentation par rapport à 2021- j'insiste, 500 % d'augmentation L'incapacité des agriculteurs à réfrigérer les plants entraînerait une chute de la production de pommes de terre. Or celle-ci est déjà réduite en raison de la crise du covid, de la multiplication des pucerons et des sécheresses de l'été 2022.

pourraient voir leur production compromise. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour venir en aide à ces producteurs de pommes de terre ? La parole est à M. le ministre.

Le Marais poitevin, zone humide de 110 000 hectares, est aménagé sur la totalité de sa surface et l'agriculture y occupe une place prépondérante. Les prairies naturelles humides constituent le principal habitat naturel à préserver.

À compter de 2023, ce dispositif doit faire l'objet d'une révision, qui nourrit l'inquiétude de l'ensemble des acteurs du Marais poitevin, et en premier lieu des agriculteurs. Recentrés sur la zone humide du Marais, des éleveurs, notamment deux-sévriens, n'auront plus accès aux De plus, la réforme entraînera des lourdeurs administratives en raison de la mise en place de l'obligation de réaliser un diagnostic d'exploitation et d'élaborer un plan de gestion pour chaque parcelle engagée. L'exploitant agricole aura également l'obligation de suivre une formation dans les deux premières années de son contrat et d'enregistrer ses pratiques au fil de l'année.

Les diminutions des montants perçus par les éleveurs auront des impacts sur la situation financière des exploitations, sur l'accélération de la diminution du nombre d'éleveurs et sur la gestion des prairies. Concrètement, les montants des indemnités par hectare vont être revus à la baisse.

mesures, adaptées à la diversité des contextes économiques, environnementaux et agronomiques des territoires- vous avez décrit les spécificités du vôtre, monsieur le sénateur. Chaque cahier des charges du catalogue est assorti d'un montant unitaire national, qui permet de compenser les surcoûts et le manque à gagner résultant de la mise en oeuvre des obligations prévues- c'est d'ailleurs le principe qui sous-tend ces mesures Ces montants ont fait l'objet d'une vérification par un organisme extérieur à l'administration, conformément à la réglementation européenne en vigueur. En particulier, concernant la nouvelle Maec relative au maintien en eau des zones basses de prairies dans les marais,

toutes les surfaces de l'exploitation peuvent faire l'objet d'un engagement dans le cadre des mesures prévues, y compris les surfaces en bandes tampons le long des cours d'eau pour lesquelles il existe une interdiction de fertilisation du fait de la conditionnalité. La baisse du montant unitaire pourra donc être compensée par une augmentation des surfaces engagées des exploitations. En outre, l'absence de rémunération de l'interdiction de fertilisation permet d'ouvrir la mesure à tout le territoire, y compris en zone vulnérable. Ces différents éléments ont fait l'objet de discussions avec les différentes parties prenantes. Il convient enfin de noter que le cumul entre la Maec relative au maintien en eau des zones basses

et numérique. Ma question porte sur la clarification du régime fiscal applicable à la solution adaptée et sécurisée de prise en charge des personnes en perte d'autonomie, qu'elles soient âgées et/ou en situation de handicap, handicap, qu'est l'accueil familial. Selon la doctrine fiscale, les personnes contraintes de recourir à l'accueil familial bénéficient du maintien d'avantages fiscaux auxquels elles auraient eu droit, le cas échéant, si elles étaient restées chez elles en ayant recours à une aide à domicile.

Or ni la loi ni la doctrine ne précisent explicitement si le recours, par un bénéficiaire, à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en oeuvre d'un séjour en accueil familial, aux côtés des conseils départementaux, ouvre droit lui aussi à un crédit d'impôt. Je souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.

de perte d'autonomie de leurs proches. Vous sollicitez en particulier une clarification publique de l'éligibilité au crédit d'impôt « services à la personne » (Cisap) des dépenses liées à ce que l'on appelle l'accueil familial. L'accueil familial permet à une personne âgée ou handicapée d'être accueillie au domicile d'une personne rémunérée pour cette prestation. La personne hébergée signe avec l'accueillant familial un contrat qui fixe les conditions matérielles, humaines et financières de l'accueil. Le coût de l'accueil comprend différentes charges supportées par l'accueillant, comme la préparation des repas ou le repassage, ainsi que la rémunération de ce dernier. Comme vous le soulignez, ces prestations entrent pleinement dans le champ du crédit d'impôt. En effet, afin de ne pas désavantager les personnes contraintes de recourir à l'accueil familial, ces dernières bénéficient du maintien des avantages fiscaux auxquels elles auraient eu droit, le cas échéant, si elles étaient restées chez elles en ayant recours à une aide à domicile. Elles sont ainsi éligibles au Cisap. Concrètement, lorsque la pièce d'habitation au sein de la famille d'accueil constitue la résidence principale ou secondaire du bénéficiaire du crédit d'impôt, la rémunération de l'accueillant ouvre droit au Cisap. La question que vous posez renvoie à une situation particulière, qui est celle des dépenses de coordination et d'intermédiation. Les activités visées peuvent être assurées par des plateformes de services à la personne, les groupements d'employeurs exclusivement dédiés aux services à la personne ou les unions et fédérations d'associations. Comme cela est confirmé dans la circulaire du 11 avril 2019 relative à la déclaration et à l'agrément des organismes de services à la personne, les dépenses engagées en vue de financer les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et à délivrer des services à la personne et qui sont rendues à la résidence du contribuable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt. Par conséquent, je vous confirme que cette règle vaut également en cas d'accueil familial. Les dépenses engagées au titre du recours à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en oeuvre de la délivrance de services à la personne éligibles au crédit d'impôt,

Novarhéna devait être un outil de « projet de territoire », lancé en grande pompe par le ministre de la transition écologique de l'époque et annoncé comme étant « la référence à l'échelle européenne en matière d'économie bas-carbone

société devait donc être « la » locomotive de la reconversion du territoire de Fessenheim. Ce sera surtout un fiasco, qui aura coûté au passage un demi-million d'euros.

Aujourd'hui, on sait que la fermeture de Fessenheim était une décision politique et idéologique, mais surtout une erreur alors que la centrale était sûre, rentable et qu'elle faisait vivre plus de 2 000 foyers. Emmanuelle Wargon, alors secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique, avait annoncé que le Gouvernement « serait au rendez-vous au moment où l'arrêt de la centrale aura vraiment un impact ». Le rendez-vous est arrivé ... Monsieur le ministre, à quoi a servi ce demi-million d'euros

a conduit à une remise en question profonde du modèle économique et social sur lequel le développement du territoire s'est appuyé ces dernières décennies. Le développement d'activités tournées vers l'industrie du futur, l'innovation, les énergies, la culture et l'agriculture constitue une réelle opportunité pour le Haut-Rhin. Conformément à son ambition, l'État s'est engagé dans un projet de territoire pour accompagner la reconversion du territoire, améliorer sa desserte et en faire un modèle de transition et d'innovation. C'est dans ce cadre que la société d'économie mixte (SEM) Novarhéna a été créée en 2019, simultanément à la signature du projet de territoire. Ce dernier a déjà donné lieu à de nombreuses concrétisations. Je pense à des projets photovoltaïques locaux et de méthanisation, à l'extension du port Colmar/Neuf-Brisach, dans lequel l'État est investisseur, ou au début du chantier d'aménagement de la zone d'activité de Novarhéna. C'est précisément au regard de l'ambition que nous avons pour le territoire de Fessenheim que la décision de dissolution de la SEM a été prise, compte tenu de la faible surface auquel elle pouvait candidater. Cette décision ne en cause le projet de territoire. En effet, de nombreux autres projets sont à l'étude. Ils traduisent notre ambition constante pour l'avenir du territoire de Fessenheim, d'abord dans le domaine des transports. Je pense à la rénovation de la ligne de fret Colmar-Volgelsheim,

le projet de technocentre porté par EDF. Ce projet, conçu par EDF et Orano, permet, vous le savez, d'envisager le renforcement d'une économie circulaire au sein de la filière nucléaire.

reconversion : c'est notre défi collectif pour le territoire de Fessenheim, emblème des enjeux territoriaux de la transition écologique. Je veux le dire ici : les perspectives économiques du territoire sont réelles et enthousiasmantes. Elles permettront au territoire de se diversifier tout en s'appuyant sur sa riche histoire dans le nucléaire. Soyez assuré, monsieur le sénateur, de la mobilisation du Gouvernement sur ce dossier.

et numérique. Monsieur le ministre, ma question porte sur les effets possibles et redoutés du système de location-gérance mis en place par le groupe Carrefour et les risques que cette externalisation fait peser sur les salariés et sur leurs droits. Dans le département des Côtes-d'Armor, Carrefour envisage de confier la gestion de son hypermarché de Langueux, près de Saint-Brieuc, à une entreprise tierce dans le cadre d'une location-gérance. Ce serait également le cas du site de Guingamp, le site de Paimpol étant déjà passé sous ce statut. À Trégueux, 230 salariés sont concernés et inquiets. Les exemples se multiplient : en 2023, la direction de Carrefour prévoit de faire passer 41 magasins, dont 16 hypermarchés, en location-gérance. La location-gérance permet au groupe Carrefour d'externaliser les salariés de ses magasins et donc de ne pas payer les salaires dans les mêmes conditions, tout en gardant la maîtrise sur l'enseigne, l'activité et les profits. Il s'agit d'un système intéressant pour les dirigeants de Carrefour et ses actionnaires, mais beaucoup moins pour les salariés. Ces derniers ne pourront plus bénéficier des avantages sociaux de l'entreprise mère, ce qui entraînera leur précarisation, car ils ne seront plus protégés par la convention collective. Alors que le groupe a présenté au mois de novembre son plan stratégique « Carrefour 2026 », qui doit notamment permettre de réaliser 4 milliards d'euros d'économies d'ici à quatre ans, Carrefour se veut rassurant en indiquant qu'aucune décision n'a encore été prise. Il rappelle que cette stratégie engagée depuis quelques années, qui consiste à passer en location-gérance des magasins déficitaires,

Cette modification est encadrée et présente des garanties pour les salariés. En cas de location-gérance, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ce contrat est utilisé par près de 2 000 entrepreneurs chaque année. À jurisprudence constante, il ressort de l'analyse de la Cour de cassation que la mise en location-gérance de magasins du groupe Carrefour n'entraînera aucune modification des éléments essentiels du contrat de travail des salariés concernés par le transfert, notamment en matière de rémunération et de conditions de travail. S'agissant du statut collectif, la location-gérance emporte la mise en cause des accords collectifs. En effet, les conventions et accords collectifs restent applicables à l'ensemble des salariés jusqu'à l'entrée en vigueur de conventions ou accords de substitution. À défaut d'accord, les dispositions conventionnelles continuent à s'appliquer pendant un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois, soit quinze mois au total. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été conclu d'accord d'adaptation ou de substitution, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. S'agissant de la convention collective de branche applicable, deux situations sont possibles. Si l'entreprise qui reprend l'activité est soumise à la même convention collective, il n'y a pas de changement pour le salarié, qui continue à en bénéficier. Si elle relève d'une convention collective différente, l'application de l'ancienne convention collective de branche des salariés transférés sera automatiquement et cessera après un délai maximum de quinze mois. Concernant la mise en location-gérance de magasins du groupe Carrefour, il est probable que l'activité reste la même. La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire devra alors continuer de s'appliquer. Il ressort ainsi que le cadre législatif existant de la location-gérance protège le droit des salariés tout en constituant une opportunité pour tous les entrepreneurs. Il n'apparaît donc pas nécessaire de modifier la législation en vigueur.

premières. Nous avons agi sur trois fronts. D'abord, en exigeant des fournisseurs qu'ils adoptent des comportements responsables. Nous avons signé une charte pour que toutes les entreprises aient une offre adaptée. Ensuite, en mobilisant l'appareil d'État pour répondre aux questions et besoins des entreprises. C'est le rôle, notamment, des conseillers départementaux à la sortie de crise.

parmi ces entreprises, celles qui sont énergo-intensives et dont la facture, après prise en compte de l'amortisseur, représente plus de 3 % de leur chiffre d'affaires, auront accès à une aide versée par la direction générale des finances publiques. C'est un nouveau soutien de l'État, qui prendra donc à sa charge environ 35 % de la hausse de la facture d'électricité.

Tous font face à des choix compliqués de réorganisation de leur production ou d'établissement de leurs prix, par exemple. Il est essentiel que les entreprises se saisissent des aides qui existent. Je vous encourage donc à diffuser la liste des conseillers départementaux à la sortie de crise aux entrepreneurs que vous rencontrez, afin que ceux-ci soient accompagnés dans cette période difficile.

Mais si ce gain est important, il n'est pas suffisant pour permettre aux exploitants d'assumer un coût d'irrigation trop élevé par rapport à leur gain de production.

l'écoute. Comme pendant la crise sanitaire, les ministres de Bercy et l'ensemble des équipes du ministère, à Paris comme dans les départements, sont mobilisés pour répondre aux inquiétudes des entreprises, adapter les aides si besoin est, regarder ce qui peut être

le site impot.gouv.fr, un ensemble de services- foire aux questions, simulateur de calcul des aides, modèles de documents -permet aux entreprises de s'informer sur les dispositifs et de trouver des renseignements précis en fonction de leur situation. Par ailleurs, un numéro vert est disponible, le 0806 000

Conscient de l'implication permanente des élus locaux, le Gouvernement a souhaité revaloriser les plafonds de ces indemnités, en portant une attention particulière aux élus locaux des petites communes, dans le cadre de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. L'article 92 de ce texte a ainsi augmenté le barème indemnitaire des maires et des adjoints de 50 dans les communes de moins de 500 habitants, de 30 % dans les communes de 500 à 999 habitants, et de 20 % dans les communes de 1 000 à 3 499 habitants. Pour accompagner cette évolution, la loi de finances pour 2020 a augmenté de 28 millions d'euros la DPEL, portant son montant total

Ciblée sur les seules communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant ne dépasse pas 125 % de la moyenne, elle s'adresse aux communes rurales les moins peuplées, dont les budgets sont les plus contraints et qui disposent donc de marges de manoeuvre réduites pour voter des indemnités à leurs maires et adjoints. Cette dotation n'avait pas été augmentée depuis 2010. Les 36 millions d'euros supplémentaires votés en 2020 sont un véritable gage de reconnaissance de l'engagement de nos élus. Par ailleurs, l'ensemble des communes sont bénéficiaires de l'augmentation de la dotation générale de fonctionnement prévue par le projet de loi de finances pour 2023, qui permettra de soutenir le financement de leurs dépenses de fonctionnement. Cette dotation sera en effet revalorisée de 320 millions d'euros, parmi lesquels 200 millions d'euros seront consacrés à l'augmentation de la dotation de solidarité rurale- dont bénéficie en 2022 la commune d'Oris-en-Rattier, à hauteur de 4 907 euros.

soulignent l'importance cruciale de leur secrétaire de mairie pour mener à bien les chantiers de leur mandat. Budget communal, documents administratifs et techniques, accueil des habitants, organisation du du conseil municipal, gestion des ressources humaines sont autant de tâches pour lesquels les secrétaires de mairie sont essentiels. Dans nos petites communes rurales, ils sont l'incarnation de la République décentralisée. Pourtant, ils sont en voie de disparition. Le déficit de reconnaissance s'est creusé d'année en année, et force est de constater que le métier a nettement perdu en attractivité et que nos élus municipaux peinent à pourvoir les postes laissés vacants, notamment à la suite de départs à la retraite. Ce sujet de préoccupation croissante n'est pas nouveau en milieu rural. Il a été soulevé dès 2021 lors du déploiement des maisons France Services. Le ministère de la transformation et de la fonction publiques d'intercommunalité (AMF) pour proposer des solutions. Le 5 octobre 2021, l'AMF a présenté 26 préconisations pour réformer le métier, qui portent entre autres sur la modification du statut, l'élargissement de l'ouverture aux contractuels ou encore la création d'un regroupement d'employeurs. Toutes ces questions liées à l'attractivité des carrières des secrétaires de mairie figuraient également parmi les chantiers de la Conférence sur les perspectives salariales de la fonction publique, qui s'est achevée en mars 2022. Quelles sont les prochaines étapes envisagées par le Gouvernement pour améliorer les conditions d'exercice de ce métier en tension ? Quel est le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre, fortement attendue sur le terrain ?

les plus rurales. Il existe déjà plusieurs outils à la main des maires pour mieux prendre en compte les conditions d'exercice de leurs fonctions, notamment pour gérer leur planning lorsque les intéressés sont employés à temps incomplet, dans les plus petites communes, et donc rattachés à plusieurs employeurs. C'est souvent le cas, et il faut continuer à accompagner au mieux ces situations pour répondre à la réalité des besoins des petites communes et permettre aux agents de bénéficier globalement d'une activité à temps plein. Pour mieux reconnaître leurs responsabilités en termes de rémunération, les maires peuvent les faire bénéficier d'un régime indemnitaire pouvant aller, pour les catégories C, jusqu'à 12 600 euros brut annuels. C'est également pour mieux valoriser et reconnaître ce métier que le Gouvernement précédent a choisi de doubler, en février 2022, la nouvelle bonification indiciaire (NBI), attribuée aux secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, ce qui représente une augmentation de plus de 70 euros par mois. Nous devons désormais aller plus loin en agissant sur le recrutement, la formation, la carrière et les parcours professionnels du métier de secrétaire de mairie. Le chantier « parcours-rémunérations » que le ministre de la transformation et de la fonction publiques lancera en janvier 2023 permettra d'avancer sur ces sujets. Au-delà des aspects statutaires, les secrétaires de mairie attendent également qu'on facilite leur quotidien et qu'on leur permette un meilleur accès aux formations, à l'information, et qu'on leur permette aussi de travailler davantage en réseau. Nous devons évidemment les aider en sens, surtout quand on sait que près de 40 % d'entre eux seront à la retraite d'ici à huit Nous devons continuer à rendre ce métier attractif. Les ministres Stanislas Guerini et Dominique Faure y travaillent activement, en lien étroit avec les employeurs territoriaux. Les propositions de l'AMF que vous évoquiez sont étudiées avec beaucoup d'attention par mes collègues, tout comme celles de l'Association des maires ruraux de France (AMRF),

montrent depuis plusieurs années une tendance au déclin démographique. Cette situation, hautement préoccupante, résulte d'une inversion de la courbe des naissances, d'un vieillissement généralisé de la population et d'une émigration massive des jeunes âgés de 18 à 35 ans- en âge de procréer, donc. Le dépeuplement est

dont vous avez rappelé l'important déficit démographique. Nous devons poursuivre nos efforts pour toujours mieux accompagner nos jeunes et les préparer aux compétences dont nos territoires ultramarins ont besoin. L'apprentissage est l'un des leviers efficaces de formation des natifs sur leurs territoires, qui garantit de plus l'adéquation aux besoins des entreprises. Pour la Guadeloupe, ce ne sont pas moins de 2 570 apprentis qui se sont formés dans une entreprise du territoire, alors qu'ils n'étaient que 175 en 2017 ! Afin de permettre l'apprentissage de tous les gestes professionnels sans recourir à de la mobilité contrainte en métropole, nous allouons annuellement au conseil régional de Guadeloupe environ 6 millions d'euros pour soutenir les investissements et le fonctionnement des centres Par ailleurs, l'État s'engage durablement aux côtés des territoires pour le développement de l'apprentissage, en maintenant une aide à l'embauche d'apprentis de 6 000 euros, qui concernera bien entendu les entreprises de Guadeloupe. La réforme que nous porterons sur le lycée professionnel s'accompagnera d'une réflexion sur la carte des formations pour ouvrir des filières davantage en adéquation avec le tissu économique du territoire et plus en cohérence avec les métiers de demain. L'État, le plan France 2030, accompagnera les collectivités dans le renouvellement des plateaux techniques et la formation des professeurs aux métiers de demain pour accélérer le processus, garantir le maintien des jeunes sur les territoires et favoriser leur insertion dans les entreprises locales. Par ailleurs, pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes, le contrat d'engagement jeune est déployé depuis le 1 mars 2022. Il vise à proposer un accompagnement adapté et personnalisé aux jeunes qui en ont besoin, avec une sécurisation financière quand cela est nécessaire. Pour 2023, il est prévu de financer 300 000 entrées en contrat d'engagement jeune par le réseau des missions locales et de Pôle emploi. Enfin, pour les jeunes les plus éloignés du service public de l'emploi, sans revenu et rencontrant des difficultés de plusieurs ordres, qu'elles soient sociales, éducatives ou de santé, des appels à projets régionaux ont été lancés et seront déployés sur l'ensemble du territoire.

Le 2 novembre, lors d'une audition au Sénat, mon collègue a clairement souligné la nécessité d'adopter un cadre plus contraignant avant les prochaines élections européennes, rappelant l'urgence de durcir nos règles, y compris pour que l'industrie chimique puisse se préparer, alors que les modifications du règlement ne prendront effet que cinq ans après la révision. Le Gouvernement est conscient du caractère essentiel de cette révision pour la santé de nos concitoyens, préoccupés par la pollution chimique, et pour la protection de l'environnement. Il connaît également les inquiétudes de certains secteurs à l'égard des modifications qui pourraient être décidées et l'importance pour ces derniers d'avoir une visibilité sur le cadre à venir. la France continuera de plaider auprès de la Commission européenne et de ses partenaires européens, comme elle le fait déjà depuis des mois, pour une révision rapide

comme sur l'ensemble du territoire national, à une crise sérieuse de l'accompagnement. Entre précarisation et manque d'offre, son département connaît une pénurie d'accompagnants 8 536 élèves présentant un handicap dans les Alpes-Maritimes, 4 434 devraient bénéficier d'un soutien humain, pour seulement 1 545 AESH en poste.

nous entamons dans quelques jours l'année 2023, des parents financent sur leurs deniers privés des AESH de temps scolaire, faute d'un meilleur accompagnement ... Quelle est aujourd'hui la position du Gouvernement sur cette question si sensible ?

même démarche s'applique pour des classes à horaires aménagés- danse, théâtre et sections sportives -, ou encore pour des classes bilingues. Ensuite, l'action du ministère de l'éducation nationale s'est portée sur la mixité au sein des lycées et des collèges. Depuis la rentrée

Madame la secrétaire d'État, permettez-moi d'attirer votre attention sur la situation des conseillers pédagogiques du premier degré qui interviennent dans l'accompagnement et la formation des enseignants et qui participent à la mise en oeuvre de la politique éducative nationale. J'ai en effet été interpellé directement par l'Association nationale des conseillers pédagogiques et autres formateurs, qui s'inquiète de l'évolution des missions de ses adhérents. Depuis plusieurs années un désintérêt grandissant pour ces fonctions. Elle s'explique par une charge de travail croissante due à une accumulation de tâches administratives, à la mise en oeuvre d'un ambitieux plan de formation nationale continue des professeurs des écoles, à l'accompagnement et à la formation des contractuels, de plus en plus nombreux, ainsi qu'à un manque d'attractivité financière du métier. Face à cette situation, les enseignants se détournent des missions de formateurs du premier degré, beaucoup invoquant leur manque de formation ou une qualité de vie au travail qui se dégrade, allant parfois jusqu'au mal-être professionnel. Il est regrettable de constater le nombre croissant de postes de conseillers pédagogiques vacants ou occupés à titre provisoire par des non-titulaires du diplôme requis. Une démarche de compensation indemnitaire a certes été engagée, mais elle n'a pas bénéficié à tous les conseillers pédagogiques.

et Paralympiques. Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur la politique gouvernementale en matière de sport-santé et bien-être. Les bénéfices des activités physiques et sportives (APS) sur la santé des Français sont documentés, démontrés et reconnus. Pratiquées à tous les âges de la vie, ces dernières participent, entre autres, à la prévention collective et individuelle des pathologies, des traumatismes et de la perte d'autonomie. La dynamique des jeux Olympiques de 2024, attribués en septembre 2017, aurait pu être le catalyseur de politiques publiques de prévention plus ambitieuses, innovantes et véritablement inclusives, qui soient en mesure de répondre aux chocs de santé publique que nous subissons. En effet, la sédentarité, accentuée par la crise sanitaire, frappe toutes les catégories d'âge, et plus sévèrement les classes populaires et les jeunes. Les temps d'exposition aux écrans explosent lorsque ceux qui sont consacrés à la pratique sportive se tassent. Cela favorise l'obésité et la mortalité prématurée. Par ailleurs, le renforcement de la place faite aux APS à l'école, du premier degré jusqu'à l'enseignement supérieur, est une impérieuse nécessité. quotidienne (APQ), consacrées dans la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, et effectives depuis la rentrée de septembre dernier, marquent une première étape. Une mission sénatoriale veillera dans les prochaines semaines à l'effectivité de leur généralisation. Enfin, le défi de la dépendance et l'objectif d'allongement de l'espérance de vie en bonne santé passeront par la réduction du nombre de chutes, ainsi que par une meilleure gestion de la baisse des capacités cardio-respiratoires et de la perte de masse musculaire. Le rôle des activités physiques thérapeutiques dites adaptées est prépondérant pour traiter certaines maladies chroniques ou faire face à la perte d'autonomie. À ce titre, faut-il aller plus loin, madame la secrétaire d'État, que le remboursement de la prescription d'activité physique adaptée (APA) et systématiser le remboursement par l'assurance maladie

que la loi du 2 mars 2022 a ouvert la prescription d'activité physique adaptée à l'ensemble des médecins et élargi le champ d'application aux personnes atteintes de maladies chroniques ou présentant des facteurs de risque, ainsi qu'aux personnes en situation de perte d'autonomie.

le Gouvernement est prêt à aller plus loin. Aussi, la ministre des sports et le ministre de la santé et de la prévention ont confié au docteur Dominique Delandre une mission visant à formuler des propositions pour accélérer le développement du sport-santé. Cette mission se penchera notamment sur les 26 expérimentations dites « article 51 de proposer aux patients une prise en charge de l'activité physique adaptée. Le bilan qui en sera réalisé permettra au Gouvernement d'envisager de nouvelles mesures dans les prochains mois. Monsieur le sénateur, vous pouvez compter sur nous pour aller plus loin. La parole

des hôpitaux ne permet pas la présence permanente des parents auprès de leur bébé hospitalisé, alors même que cette présence est prévue dans la nouvelle charte du nouveau-né hospitalisé, établie par le Gouvernement en novembre 2021.

par la carence de médecins, de pédiatres spécialisés et de personnel paramédical en puériculture, toute organisation nouvelle permettant de soulager ces services serait opportune et bienvenue.

La proposition, déjà très élaborée et affinée par l'équipe du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, a fait l'objet d'un courrier adressé au ministre de la santé et de la prévention, qui est resté à ce jour sans réponse. Devant l'importance de cette proposition, j'ai également saisi les services de Mme la Première ministre et j'en ai fait l'objet de la question de ce jour. Le sud de la France étant déjà peu pourvu en services de néonatalogie au regard de sa population, madame la ministre, de prendre en considération cette proposition d'équipe mobile, en raison des avantages considérables que cette alternative à l'hospitalisation traditionnelle offrirait aux familles.

En Paca, deux établissements, dont le centre hospitalier intercommunal Sainte-Musse à Toulon, ont exprimé leur souhait de développer des équipes mobiles de néonatalogie, en déposant des projets de qualité conformes aux attendus réglementaires. La dimension territoriale affirmée du projet et les synergies entre la ville et l'hôpital constituent des atouts qui ont été soulignés lors de l'analyse des dossiers. Le service de néonatalogie du centre hospitalier de Toulon est un acteur incontournable à l'échelle régionale. Situé entre les deux métropoles de Marseille et de Nice, il répond aux besoins de l'ensemble du département du Var et, par extension, des départements limitrophes. Son équipe médicale et paramédicale possède les savoir-faire pour accueillir, prendre en charge et accompagner les nouveau-nés et leurs parents pendant l'hospitalisation et au décours. Par ailleurs, il s'agit d'une des équipes pilotes en soins de développement. Ces acquis seront transférables dans le cadre du projet d'équipe mobile. Au-delà de la qualité intrinsèque du dossier, l'ARS a souligné le consensus et l'engagement collectif autour de cette expérimentation, qui bénéficie d'un fort soutien de la direction de l'établissement comme des représentants des usagers. Par conséquent, le ministère a sélectionné ce projet parmi ceux qui feront partie de l'expérimentation et qui seront annoncés dans un arrêté à paraître prochainement.

-le traitement des dossiers administratifs de santé des citoyens italiens, ne prend plus en charge les consultations en faveur de ces derniers. Ainsi, une partie non négligeable des consultations qui sont réalisées au centre hospitalier des Escartons, à Briançon, soit à quelques kilomètres de la frontière italienne, n'est plus remboursée. Cela a pour conséquence un manque à gagner de plus de 2,5 millions d'euros

% en chirurgie - et 25 % des professionnels médicaux et praticiens de cet établissement sont italiens, majoritairement piémontais. L'absence d'accord transfrontalier en matière de sécurité sociale risque, en définitive, de réduire la fréquentation de l'établissement et de favoriser le départ des professionnels de santé qui ne pourraient plus organiser la continuité des soins. Car oui, l'Italie est le seul État frontalier de l'Hexagone avec lequel nous n'avons pas, à ce jour, d'accord d'une telle nature ! Mon interrogation est donc double, madame la ministre. Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour préserver transitoirement la situation financière du centre hospitalier des Escartons

Quelles sont donc les initiatives prises par le Gouvernement pour achever la mise en oeuvre et la ratification d'un tel accord transfrontalier franco-italien de prise en charge de la patientèle italienne ?

déléguée. Monsieur le sénateur, attentifs à la situation du centre hospitalier de Briançon, les services du ministère de la santé ont pris contact avec les différents acteurs impliqués, notamment la CPAM et l'ARS, afin d'apporter non seulement une réponse de court terme, mais également une solution pérenne aux patients frontaliers. Des actions seront engagées pour traiter les dossiers litigieux dans les jours à venir. Aussi, le risque de départ des professionnels de santé italiens est un sujet pris en considération dans la recherche de solutions à court et moyen termes. À moyen et long termes, dans la continuité des travaux engagés depuis 2021, les autorités françaises sont favorables à la mise en place d'une coopération sanitaire avec l'Italie. Les services du ministère, les ARS, ainsi que notre ambassade à Rome, ont travaillé à un projet d'accord de coopération sanitaire transfrontalier franco-italien, qui s'inscrit pleinement dans le cadre du traité du Quirinal, qui devrait entrer en vigueur au début de 2023. Ce projet de coopération, qui vise notamment à encadrer juridiquement et à faciliter les soins des populations dans les territoires enclavés ou mal desservis, a quant à lui été transmis aux autorités de santé italiennes au début du mois de juillet 2022. Il est depuis à l'étude. Nos services Nos services demeurent en contact régulier avec leurs interlocuteurs italiens pour souligner l'attachement de la France à la signature de cet accord. La nouvelle équipe ministérielle italienne étant désormais installée, notre ambassade a prévu d'entamer une nouvelle démarche auprès de nos homologues.

L'utilisation exponentielle des antibiotiques, en santé tant humaine qu'animale, est la cause principale de ce phénomène, et nous nous dirigeons probablement vers des impasses thérapeutiques dans le traitement de nombreuses maladies infectieuses. L'antibiorésistance est un problème mondial, qui pourrait devenir Cette réalité est encore trop méconnue du grand public, malgré une sensibilisation régulière de nos concitoyens et une mortalité attribuable à l'antibiorésistance en France estimée à 5 500 décès.

Les antibiotiques, c'est pas automatique » : nous nous en souvenons tous. La prévention de l'antibiorésistance appelle un engagement fort des pouvoirs publics, intégrant la santé animale et des écosystèmes, dans une approche globale. La feuille de route interministérielle dédiée, publiée en 2016, est ainsi en cours d'actualisation. Des progrès sont à souligner : les prescriptions d'antibiotiques en ville ont baissé de 20 % entre 2009 et 2019 et la consommation en établissement connaît une tendance baissière. Pour autant, notre consommation d'antibiotiques reste trois fois supérieure à celle des plus faibles consommateurs européens et les niveaux d'antibiorésistance sont toujours préoccupants en France. Dans le sillage des plans précédents, le ministère de la santé a publié en février 2022 sa stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance, avec une vision renouvelée et ambitieuse. Elle repose sur deux piliers complémentaires : le bon usage des antibiotiques et les actions de prévention et de contrôle des infections. Ne pas tomber malade réduit en effet le recours à l'antibiothérapie et donc l'antibiorésistance. Les professionnels et citoyens y sont fortement associés, par une formation renforcée et des campagnes de communication dédiées. Ces objectifs sont pilotés au niveau régional par les ARS, appuyées par des structures locales et des équipes mobiles. Ce maillage territorial fin est une spécificité française. La France travaille également au développement de nouveaux produits luttant contre l'antibiorésistance, en complément d'une prévention renforcée. Enfin, il convient de souligner le vif engagement international de la France sur ces thématiques, notamment à l'échelle européenne.

Les coûts engendrés par l'antibiorésistance se chiffrent en centaines de milliards d'euros à l'échelle mondiale et, vous l'aurez compris, l'urgence est là. « Les antibiotiques, c'est pas automatique »- la formule est en effet dans tous les esprits -, mais ce n'est pas magique non plus. Il faut un engagement de la part, à la fois, des prescripteurs et des pharmaciens. La bonne observance thérapeutique est évidemment

Si la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a bien prévu, dans son article 39, la prise en charge par l'assurance maladie des dispositifs médicaux remis en bon état d'usage, le décret d'application n'a toujours pas été publié. Dans un contexte de crise économique et sociale, où les actions pour lutter contre l'inflation semblent être une priorité pour le Gouvernement, il est étonnant que ce décret n'ait toujours pas entériné la mesure votée en 2019.

l'accès aux aides techniques et d'accélérer le déploiement de l'économie circulaire en matière de matériel médical. Cette réforme d'envergure nécessite des discussions approfondies avec les nombreux acteurs impliqués. Les échanges se structurent autour de plusieurs textes qui sont nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi Le décret d'application est notamment couplé à une norme en cours d'élaboration. Travaillée avec toutes les parties prenantes au cours de l'année 2022, celle-ci permettra de définir les activités et les responsabilités des acteurs de la remise en bon état d'usage. Ces travaux importants serviront de socle au développement de cette activité. Il convient donc de prendre le temps nécessaire. En pratique, les services du ministère m'ont remis un projet de décret finalisé, que nous allons soumettre pour avis au Conseil d'État afin de permettre une publication au deuxième trimestre 2023. La norme que j'ai évoquée servira également de socle à l'homologation des centres qui réaliseront les activités de remise en bon état d'usage. Plus largement, le déploiement de l'économie circulaire est un élément important dans la réalisation de l'ambition gouvernementale d'amélioration des conditions d'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap. Pour renforcer encore notre ambition, nous prévoyons de reprendre les négociations tarifaires avec les industriels et distributeurs de matériel médical, afin de faire aboutir la réforme de la prise en charge, entamée voilà un peu plus d'un an.

rétribué 2,32 euros : ce système pénalise les territoires ruraux, où la garde est bien souvent éloignée du lieu de prise en charge du patient et des centres hospitaliers. Deuxièmement, l'instauration d'un nouveau mode de calcul le revenu minimum garanti (RMG), qui est de 64 euros de l'heure ou de 768 euros pour une garde de douze heures, est elle aussi pénalisante. En effet, il faut déduire de ce RMG

L'indemnité de garde de 346 euros est remplacée par la notion de revenu minimum garanti : ce RMG a été mis en place afin d'inciter les transporteurs à effectuer des gardes, en particulier dans les secteurs ruraux où il y a peu d'interventions. Dans le cas où le transporteur n'assure pas suffisamment de trajets pour couvrir ses charges, un complément est versé. Les interventions non suivies de transport sont également prises en charge, à hauteur de 80 euros. D'un point de vue organisationnel, la réforme permet d'assurer une garde ambulancière sur l'ensemble des plages horaires ; mais cette répartition, par horaire et par secteur, est modulée dans chaque territoire selon les besoins d'intervention locaux. Une logique de seuil a servi de base à la définition du positionnement des moyens de garde par période.

Le ministère est très attentif aux remontées du terrain quant à l'application de cette réforme ; pour accomplir de nombreux déplacements, je sais très bien que c'est un véritable enjeu. Le bilan financier relatif au circuit de paiement effectué sera communiqué en fin d'année et un bilan organisationnel est prévu pour le premier trimestre 2023. Des discussions pourront être ouvertes en vue d'éventuels ajustements.

La question du « bien vieillir » et de l'autonomie dans notre territoire est une préoccupation réelle. À ce titre, le département de la Haute-Loire et les acteurs locaux se mobilisent au bénéfice des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, dans le cadre du déploiement d'habitats inclusifs.

Ces lieux de vie constituent une réponse prometteuse pour sortir du dilemme vécu par les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, lorsque la vie collective en établissement n'est ni souhaitée ni nécessaire et lorsque la vie chez soi, comme avant, n'est plus possible. Le vieillissement et l'autonomie sont des problématiques majeures pour les territoires ruraux. Il est nécessaire d'opter pour une approche pragmatique, mêlant le public et le privé : il est donc indispensable que l'État puisse envisager de nouveaux dispositifs afin de valoriser ces habitats.

ministre déléguée. Monsieur le sénateur, vous avez raison de rappeler l'importance de l'aide à la vie partagée. L'AVP vise à permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap de financer les coûts d'une vie partagée dans l'habitat inclusif. Elle contribue ainsi pleinement à favoriser le libre choix du lieu de vie.

%. On anticipe que le financement par la CNSA restera stable jusqu'en 2025, autour de 45 millions d'euros par an, et qu'il augmentera avec la croissance de l'habitat inclusif. Le développement de ce mode d'hébergement repose en effet sur une politique incitative régulièrement discutée entre la CNSA et les conseils 96 départements auront inscrit l'AVP dans leur règlement départemental d'aide sociale et établi leur programme d'ici à la fin de l'année. Au-delà de ce dispositif, c'est bien un continuum de solutions que nous mettons en place. La mise en oeuvre de MaPrimeAdapt'permettra aux personnes aux revenus modestes d'aménager leur logement aux contraintes liées à l'âge ou au handicap. En parallèle, la prochaine Conférence nationale du handicap permettra de faire évoluer l'offre médico-sociale pour toujours mieux répondre aux attentes des personnes.

premiers jours de la vie et en formulant le souhait que la France investisse dans un programme d'accompagnement des parents, il manque en France 230 000 places de crèche, en plus des 446 000 existantes. Si notre pays a pu s'enorgueillir d'un système de la petite enfance performant, il est désormais en perte de vitesse face à ses voisins européens : aujourd'hui, 40 % des enfants n'ont aucune solution d'accueil.

Certes, le Président de la République et la Première ministre ont annoncé la formation de 100 000 nouveaux professionnels d'ici à 2027 ; mais encore faut-il trouver des candidats La profession n'attire plus, en raison des conditions de travail, des niveaux de salaires trop bas, de l'absentéisme non remplacé, du manque de moyens ou encore du manque de reconnaissance. Or elle

C'est l'ambition du futur service public de la petite enfance, au sujet duquel le ministre Jean-Christophe Combe a annoncé, le 21 novembre dernier, le lancement d'une grande concertation dans le cadre du

ou encore sur les salaires. Dès le mois de juillet dernier, mon collègue Jean-Christophe Combe a débloqué 2,5 millions d'euros pour créer un observatoire de la qualité de vie au travail et organiser une campagne de promotion de ces métiers. Le 22 septembre, il a confirmé que l'État accompagnerait des revalorisations salariales, sous réserve que soit défini un socle social commun pour ces métiers ; à la demande des partenaires sociaux, le Gouvernement a saisi l'inspection générale des

la mise en place progressive de la zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) est un véritable casse-tête pour les 100 000 sociétés des secteurs du bâtiment, des travaux publics et du transport routier qui exercent leur activité au sein de la métropole. sont déjà lourdement frappées par les restrictions d'accès aux communes situées dans le périmètre de l'autoroute A86. Elles le seront plus encore par la limitation de circulation qui s'appliquera aux véhicules classés Crit'Air 3 à partir du 1 juillet 2023, comme l'a décidé le conseil de la métropole du Grand Paris. Comment desservir les chantiers en cours, assurer les livraisons ou répondre à des marchés avec des véhicules ne correspondant plus aux critères exigés ? Ces entrepreneurs s'estiment d'autant plus pénalisés que les aides de l'État, même cumulées à celles de la région et de la Ville de Paris, sont nettement insuffisantes pour le renouvellement de leurs flottes et que les offres de véhicules à faibles émissions sont inexistantes chez les constructeurs. C'est un véritable mur écologique et économique qui se dresse devant ces entreprises.

mes questions sont les suivantes : allez-vous entendre la voix des chefs d'entreprise, qui vous demandent d'agir avec souplesse et pragmatisme ? Envisagez-vous de revoir, avec leurs organisations représentatives, le calendrier de déploiement de la ZFE d'Île-de-France, afin de tenir compte des évolutions technologiques en cours

beaucoup avec lui sur ce sujet. La zone à faibles émissions mobilité fait partie des outils à la main des collectivités territoriales pour améliorer la qualité de l'air. Ces dernières définissent le périmètre d'application des ZFE, les critères et les échéances retenus. Les étapes de concertation et d'information permettent de prendre en compte les contraintes de l'ensemble des acteurs, en adaptant les horaires de restriction ou en instituant des dérogations ciblées en complément des exemptions prévues à l'échelle nationale.

Madame la ministre, comme vous le savez, dans les facultés de droit et de sciences politiques, la sélection de nos étudiants en master intervient, depuis la rentrée de septembre 2020, dès le master 1. Cette réforme est bénéfique pour les étudiants qui, dans l'ancien système, seraient passés en master 1 sans obtenir un master 2.

L'étudiant qui n'avait pas été retenu, malgré l'obtention de son master 1, devait trouver un master 2 loin de chez lui, accepter un master dans une spécialité qui n'était pas la sienne ou tout simplement abandonner l'université. Certes, avec la sélection, nous pouvons nous réjouir que les étudiants admis en master 1 aillent automatiquement en master 2 après validation de leur quatrième année. Mais ce système a aussi ses travers. C'est une réforme qui touche principalement les facultés de droit. Il faut bien avoir à l'esprit que, dans cette discipline, les étudiants choisissent aussi la voie des concours.

Ainsi, ma question est la suivante : que compte faire le Gouvernement pour remédier à cette conséquence négative de la réforme des masters ? La parole ministre déléguée. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser ma collègue Sylvie Retailleau, en déplacement en Guyane. La réforme instituée par la loi du 23 décembre 2016 a adapté le deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat conformément au processus de Bologne. Il s'agissait d'harmoniser les systèmes nationaux européens d'enseignement pour permettre une reconnaissance des diplômes nationaux dans tout l'espace européen d'enseignement supérieur. L'objectif permettre à chaque étudiant inscrit en première année de master d'achever son cursus sans subir de sélection entre la première et la seconde année ; et offrir à chaque titulaire du diplôme national de licence une poursuite d'étude, notamment le dispositif de saisine du recteur.